conformément à la décision de la conférence des présidents réunie le 1 décembre dernier. J'invite par ailleurs chacune et chacun à respecter les gestes barrières.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'eau, c'est la vie ! Elle est une ressource essentielle et stratégique pour notre planète comme pour notre pays. Je me réjouis donc que notre groupe Les Républicains ait demandé l'inscription de ce débat

l'eau. Avant d'aborder la partie « problèmes, attentes et recommandations », permettez-moi de revenir très brièvement sur la construction des agences de l'eau. pollution a consacré une nouvelle organisation de la politique publique de l'eau, fondée sur une gestion décentralisée en bassins versants, sur de grands principes permettant, à la fois, de lutter contre la pollution- en vertu du principe du pollueur-payeur -et de concilier les besoins en eau pour les collectivités, l'agriculture et l'industrie. L'objectif était de mettre en place une politique profondément décentralisée, respectant l'un des principes clés de la gestion environnementale : la subsidiarité. Avons-nous atteint cet objectif ? Poser la question, c'est y répondre ... Un premier problème doit être mis en avant. Il concerne l'absence de visibilité, et surtout la complexité du fonctionnement de ces agences.

et le préfet coordonnateur de bassin qui représente l'État au niveau de ces instances pour surveiller et coordonner l'action des bassins. Je rappelle également la création, au niveau national, du Comité national de l'eau (CNE), qui donne un avis consultatif sur les actions engagées.

Aux côtés des acteurs présents parce qu'ils ont été élus, on trouve une palanquée d'acteurs nommés- experts, associations, bientôt conseil scientifique -, qui n'aident pas à la compréhension du fonctionnement des agences de l'eau mais qui, n'ayons pas peur de le dire ! -sèment le doute sur la capacité des élus, des collectivités, des chambres consulaires, des utilisateurs et des usagers à gérer la politique de l'eau, mettant en cause leur légitimité. Une simplification du labyrinthe s'impose donc. Le deuxième problème concerne le financement des agences de l'eau et l'étendue des leurs missions, un ensemble qui pousse au non-respect d'un principe fondateur selon lequel « l'eau paye l'eau ». Comment en sommes-nous arrivés à cette situation de non-respect dudit principe ? Cela a commencé en 2010 par la politique de l'ancienne ministre de l'environnement, Dominique Voynet, qui avait mis en place tout un système visant à siphonner les excédents des agences de l'eau pour abonder le budget de l'État.

en 2018, l'abaissement du plafond de recettes des agences de l'eau, dit « plafond mordant », qui a également poussé les comités de bassin à réduire la fiscalité de l'eau et a entraîné une forte baisse des moyens alloués aux politiques des agences, notamment celles visant à venir en aide aux projets des collectivités territoriales. Notons que ces ponctions se faisaient au moment où l'on demandait aux collectivités locales de se mettre aux normes pour leur assainissement collectif, et en outre d'élargir leur domaine d'action la gestion Enfin, comment ne pas évoquer l'étendue des prérogatives des agences de l'eau ? Nous savons qu'elles sont passées de la gestion de ce que l'on appelle « le petit cycle de l'eau »- eau potable et assainissement -à celle des « grands cycle de l'eau lesquels comprennent les milieux aquatiques, le littoral, l'agriculture et la biodiversité ... Le problème est survenu avec la création de l'Office français de la biodiversité Selon les dernières données, 80 % du financement de l'OFB sont assurés par les redevances gérées par les agences de l'eau, ou au titre du littoral. Comment, dans ces conditions, assurer le principe fondateur « l'eau paye l'eau » Nous avions pourtant indiqué à maintes reprises, au Sénat, lors de la création de l'OFB, que cette instance allait poser des problèmes financiers aux agences. Comme c'est souvent le cas, nous avions tort d'avoir raison trop tôt ! Pour résumer, le message que l'État adresse aux agences est le suivant : « Faites plus avec beaucoup moins, et surtout débrouillez-vous

quand la seconde ne perçoit que 376 millions d'euros, soit un différentiel de 309 millions, et ce, alors que l'agence Loire-Bretagne regroupe deux fois plus de territoires. J'en viens à la péréquation au bénéfice des territoires ruraux. Ces derniers sont producteurs de « services environnementaux » importants dans le domaine de l'eau et de la biodiversité. Si le dispositif actuel de péréquation permet une redistribution des villes vers les campagnes, de l'aval du bassin vers l'amont, du littoral vers l'intérieur, il faut réfléchir à une évolution plus large afin de véritablement rémunérer les services environnementaux rendus par les espaces ruraux.

Nous croyions l'avoir réglé, mais le dérèglement climatique et l'arrivée massive dans les instances des adeptes du « frein à main » des projets viennent bouleverser nos certitudes. Cela nous impose de revoir ou de diversifier nos outils, qu'il s'agisse : des modalités d'intervention, de planification, de gouvernance et de décomplexification ; de la sécurisation des quantités de l'eau, élément stratégique qui passe par la simplification des procédures de retenues collinaires de la diversification des ressources financières pour faire face à l'élargissement du périmètre d'intervention des agences de l'eau en matière de biodiversité et de milieu marin ; de la péréquation et de la répartition entre les bassins des moyens disponibles, en fonction des objectifs à atteindre et de la place des territoires ruraux.

sur les agences de l'eau, passées, présentes et à venir. Les agences de l'eau sont au coeur de notre politique d'intervention pour l'eau et la biodiversité dans un contexte, que vous

d'une première séquence des Assises de l'eau portant sur la rénovation de nos dispositifs d'assainissement et d'eau potable. En 2019, une deuxième séquence des Assises de l'eau a été consacrée à l'adaptation au changement climatique et à la gestion globale de la ressource.

Aujourd'hui, toutes les collectivités le savent et s'y engagent. Les six agences de l'eau, établissements publics de l'État présents sur le territoire métropolitain, jouent

à l'environnement- prélèvements excessifs sur la ressource ; pollutions ponctuelles et diffuses dues aux rejets d'eaux usées domestiques et industrielles, ou encore aux rejets azotés ou phytosanitaires. Ces recettes permettent

marins. Conformément au souhait du Gouvernement, les agences de l'eau ont ainsi accentué l'accompagnement des projets en faveur de la gestion du grand cycle de l'eau, de la qualité des milieux aquatiques et de l'adaptation rendue nécessaire par le changement climatique.

Nous sommes au rendez-vous, puisque le 30 juin 2021, les agences avaient déjà octroyé plus de 700 millions d'euros, depuis 2019, aux collectivités rurales pour les aider à renouveler leurs installations d'eau potable et d'assainissement.

nous avons stoppé la baisse des effectifs dans les agences de l'eau. C'était une nécessité, car celles-ci ont largement participé à l'effort de maîtrise des effectifs parmi les opérateurs de l'État. Nous avons mis fin à ces baisses pour permettre aux agences de l'eau de répondre à l'élargissement de leurs missions et à leur montée en puissance.

nous savons tous que le changement climatique est l'un des enjeux majeurs de la politique de l'eau, et que les agences de l'eau ont un rôle prépondérant à jouer pour réduire les pollutions de l'eau de toutes origines, protéger les ressources en eau et lutter contre l'érosion de la biodiversité.

Les agences de l'eau sont résolument engagées dans le cadre du plan de relance. Sur les 250 millions d'euros d'aides allouées à des projets portant notamment sur la mise aux normes des stations de traitement des eaux usées et la rénovation des réseaux d'assainissement, plus de 16 millions d'euros concernent directement l'agence de l'eau Artois-Picardie. je me réjouis moi aussi bien évidemment que les effectifs des agences soient maintenus cette année, après des années de baisse historique, je souhaiterais que vous nous confirmiez que les engagements pris lors de l'annonce du plan national de gestion durable des eaux pluviales permettront réellement à l'agence Artois-Picardie de mener ses missions dans le département du Nord,

entre 2010 et 2021. Depuis 2018, les ponctions régulières sur leurs ressources et l'existence d'un plafond mordant ont limité leurs capacités opérationnelles. Pour les années 2019-2024, le budget des onzièmes programmes pluriannuels d'intervention a enregistré un recul de près d'un milliard d'euros par rapport aux précédents programmes. Parallèlement, la réforme sur les redevances perçues par les agences, qui devait être inscrite dans le projet de loi de finances pour 2022 et qui a suscité des inquiétudes l'été dernier, a été ajournée. La question de la capacité des agences de l'eau à accompagner les collectivités territoriales et les acteurs locaux dans leurs projets en matière de gestion de l'eau se pose désormais. Alors que ces agences jouent un rôle déterminant, tant dans la bonne mise en oeuvre des politiques de préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques que dans la performance des services et la maîtrise des coûts, il est urgent de trouver des stratégies de financement pertinentes et de tracer une orientation budgétaire à long terme. Nous devons aussi nous prémunir contre toute remise en question de leurs missions historiques qui serait opérée selon des calculs purement comptables. Je pense au dossier de l'assainissement non collectif, qui n'a pas été retenu parmi les priorités ministérielles en matière d'intervention des agences de l'eau pour la période 2019-2024. Dans les territoires, cela se traduit par des difficultés importantes, tandis que les aides sont de plus en plus rares pour la mise aux normes des installations et que les maires ou les présidents d'intercommunalités se retrouvent démunis face à leurs habitants.

Comment comptez-vous assurer une capacité de financement permettant aux agences de faire face à ces enjeux, notamment dans les bassins très ruraux à faible potentiel fiscal ? Comment faire jouer davantage la solidarité nationale et comment réviser le plafond des agences à la hausse afin de sécuriser leurs interventions face au changement climatique ?

L'adaptation au changement climatique préoccupe l'ensemble des usagers de l'eau. Le débit moyen annuel des rivières devrait baisser de 10 % à 40 % au cours des prochaines décennies, ce qui conduira inévitablement à des conflits d'usage. La question du partage d'une ressource dont la quantité et la qualité sont menacées implique donc de définir des orientations fortes à l'échelle nationale. En dépit de cet objectif commun, nous constatons des divergences d'application des politiques publiques menées par les agences de l'eau, selon les bassins versants.

la création de retenues collinaires, qui permettent de récupérer les excédents d'eau en période hivernale ou en période de crue pour les restituer en période de stress hydrique, ne fait pas l'objet d'une même doctrine et ne bénéficie donc pas des mêmes financements ici ou là, ce qui accentue les tensions locales. Après les assises de l'eau de 2018 et 2019, l'initiative du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique était bienvenue : elle doit permettre, grâce au dialogue et à la concertation, de construire des solutions pour l'avenir dans un cadre apaisé, l'agriculture étant particulièrement vulnérable.

innovantes et pragmatiques, libres de tout raisonnement dogmatique.

nous sommes confrontés au problème de la pollution de la Moselle par les rejets de chlorures nocifs des soudières de la vallée de la Meurthe. À ce titre, les gouvernements successifs n'ont strictement rien fait. Ils ont même cautionné ces pollueurs scandaleux, puisque, chaque fois que de l'argent public a été investi pour écrêter les pics de pollution en période d'étiage, c'est-à-dire en été, les soudières en ont profité pour augmenter leur pollution. Actuellement, ces entreprises rejettent deux fois plus de chlorures nocifs dans la Moselle

à l'horizon de 2050. La température de l'eau frise alors les 30 degrés. Aux sécheresses de plus en plus fréquentes et sévères s'ajoute l'augmentation de la distribution d'eau à Toulouse et à Bordeaux, métropoles très attractives qui accueillent chacune quelque 15 000 habitants de plus chaque année. Nous sommes ainsi confrontés à une équation bien difficile à résoudre et les enjeux, déjà nombreux, ne cessent de se multiplier. Si le réchauffement climatique s'installe petit à petit dans ce qui s'apparente à un voyage sans retour, nous devons aussi faire face au constat alarmant d'une accumulation de micropolluants dans les eaux de nos rivières

et il est à craindre que l'augmentation des moyens nécessaires ne pèse sur nos concitoyens, comme c'est le cas aujourd'hui. En effet, plus de 70 % des revenus perçus par les agences de l'eau viennent des particuliers. La reconquête et le bon état de nos masses d'eau exigent non seulement une organisation locale aussi, bien entendu, des moyens financiers et humains à la hauteur des enjeux. La première stratégie des agences de l'eau est de réussir à préserver ce bien commun essentiel. Les comités de bassin sont des lieux de dialogue et d'équilibre entre personnes qualifiées, et associations. Cet esprit de concertation et le caractère décentralisé de cette gouvernance sont les mieux à même de répondre aux situations locales. entendez-vous poursuivre le gel de la baisse des effectifs de ces agences au-delà de 2022 ? Comment comptez-vous assurer une adaptation responsable au dérèglement climatique et aux pollutions diffuses ?

L'article L. 210-1 du code de l'environnement définit l'eau comme faisant « partie du patrimoine commun de la Nation ». Les agences de l'eau ont été créées en 1964 pour favoriser la solidarité territoriale et financer non seulement le petit cycle de l'eau, mais encore la prévention, en amont.

Par ailleurs, face aux défis climatiques qui seront, demain, plus importants et plus nombreux qu'hier pour les agences de l'eau, le principe de plafond mordant, introduit par la loi de finances pour 2018, a-t-il encore du sens ? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice

Ce projet ambitieux, de 17 millions d'euros sur dix ans, est un programme global de production indirecte d'eau potable à partir d'eaux usées. Après traitement, il serait question non plus de les rejeter à la mer, mais de les réinjecter dans le circuit de l'eau potable à l'issue d'un processus comprenant une unité d'affinage et une zone

L'agence de l'eau accompagne Vendée Eau pour la première phase du projet, à hauteur de 4 millions d'euros sur les 9 millions engagés à ce jour, mais elle refuse d'envisager un soutien à l'intégralité du projet. Ainsi, la canalisation, la zone végétalisée et les études d'impact indispensables à la réalisation de ce projet ne seraient pas éligibles à une aide, ce qui risque de compromettre l'expérimentation de la démonstration qui doit faire avancer la réglementation, sauf à s'orienter vers un financement privé. Madame la secrétaire d'État, pouvons-nous raisonnablement confier à des sociétés privées le soin d'offrir une réponse à la ressource en eau, alors qu'un organisme d'État est censé s'y consacrer ? Pouvez-vous enfin vous engager à financer ce projet ? La parole

ce projet. Les prochaines phases, qui concernent la canalisation et les ouvrages associés, la zone de transition et les études et bilans, sont estimées à 13 millions d'euros par le syndicat départemental. Nous sommes donc à la recherche de financements complémentaires dans le cadre d'un tour de table. La vision globale des prochaines étapes du projet doit inclure la démonstration de son caractère reconductible. L'ensemble

Depuis le début de mon mandat, je suis régulièrement interpellée par les maires de petites communes qui éprouvent de plus en plus de difficultés dans leurs rapports avec l'agence de l'eau de notre bassin. Pour ces collectivités territoriales, la mise aux normes de l'assainissement, imposée par les mêmes agences de l'eau ou par les établissements

Le programme des agences de 2014 abandonnait le financement du collectif au profit du non-collectif. De nombreuses communes ont alors commandé des études dans l'espoir de bénéficier des subventions des agences. Mais le onzième programme, entré en vigueur en 2019, ne subventionne plus le non-collectif. Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation des études, des délais d'instruction et des fréquents changements des zonages déterminés par les agences, les communes n'ont tout simplement pas pu bénéficier des subventions du dixième programme.

Madame la secrétaire d'État, alors que les fonds du plan de relance sont censés favoriser les travaux de mise aux normes environnementales de l'assainissement, les communes rurales ont besoin de savoir si le non-collectif fait partie des priorités de l'État. Dans l'affirmative, comment mobiliser enfin des subventions à leur profit

bien au-delà de leurs compétences propres : Agence française pour la biodiversité (AFB), parcs nationaux et j'en passe. Plutôt que d'accorder à ces opérateurs des crédits propres, le Gouvernement puise dans le budget des agences de l'eau, lui-même constitué de redevances payées par tous les usagers. de l'eau financent actuellement près de la moitié des politiques de la biodiversité. Mais cela ne s'arrête pas là : vous avez institué un plafond mordant, autrement dit un seuil, fixé à 2,1 milliards d'euros en 2019, au-delà duquel les recettes perçues par les agences sont directement reversées au budget de l'État.

Ledit rapport rappelle que les agences sont des acteurs essentiels de la préservation de l'eau : elles mènent ou financent des actions de dépollution, d'entretien des réseaux et de restauration des rivières.

multiplication des inondations et des sécheresses, raréfaction des ressources en eau, élévation du niveau de la mer en raison du dérèglement climatique, etc. Ce sont là autant de sujets qui vont nécessiter des actions de grande ampleur. D'ici à la fin du siècle, les agences de l'eau prévoient une baisse de 10 % à 50 % du débit d'étiage des grands fleuves et de 10 % à 30 % des nappes phréatiques, ce qui entraînera une plus grande concentration des polluants dans les rivières. des polluants dans les rivières. En organisant, par le biais du plafond mordant, l'attrition des finances des agences de l'eau, ne nous éloignons-nous pas du modèle décentralisé de gestion de l'eau par les agences et les comités de bassin et, de fait, du principe selon lequel l'eau paye l'eau ?

des métropoles (Maptam) a créé une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, la Gemapi, attribuée exclusivement aux communes. Le but est d'assurer une approche plus globale, à l'échelle d'un bassin versant, de la qualité de l'eau et de la préservation des zones humides.

en dehors de leur champ de compétence, mais surtout en contradiction avec les priorités fixées par les syndicats mixtes compétents, ce qui suscite des tensions et fait peser des contraintes sur les autres membres du syndicat.

La situation de conflit d'intérêts n'est pas établie, d'autant qu'aucun élu de la communauté de communes n'est membre des instances de l'eau. En tout état de cause, les personnes susceptibles d'être en situation de conflit d'intérêts ne participent ni aux débats ni aux votes. Le ministère a été particulièrement vigilant au respect des règles de déontologie dans l'attribution de ces aides publiques. À ce titre, les administrateurs des agences de l'eau sont soumis au respect d'une charte de déontologie dont les exigences sont définies par un arrêté ministériel du 5 février 2021.

Las, par endroits, ce n'est pas encore une réalité. Afin d'organiser le plus efficacement possible la compétence Gemapi en sécurisant les structures existantes, il vous faudrait lever certaines imprécisions, notamment quant aux limites de compétences et aux responsabilités liées des agences de l'eau.

Pierre angulaire de notre politique nationale de l'eau, la loi de 1964 a institué les six agences que nous connaissons. Le principe fondateur du financement de ce service public était alors clairement défini : l'eau paye l'eau. Or les élus locaux constatent aujourd'hui que ce principe est plus que jamais menacé. J'en donnerai deux exemples. Le plus criant concerne les financements nécessaires au renouvellement des réseaux : beaucoup de petites et moyennes communes ne parviennent pas à obtenir les aides suffisantes

comment expliquer au maire d'une petite commune de Beauce que l'agence Loire-Bretagne concentre ses financements sur la prévention et non sur la réduction de la teneur en nitrate de l'eau potable, alors que la France est mise en demeure

car il s'agit d'un enjeu majeur pour nos élus locaux. Je ne suis pas certain que vous ayez pris la pleine mesure de l'urgence et de la difficulté de leur situation. Garantir l'usage économe d'une eau potable de bonne qualité, à un coût raisonnable, est peut-être le premier des combats écologiques.

le manque de cohérence et de lisibilité du projet, la vision dogmatique du changement climatique, sous le seul angle de la pénurie d'eau, et l'absence de possibilités de stockage ou de création de ressources.

est suspendue. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d'accueil sur le territoire français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

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l'histoire des harkis, c'est l'histoire de France. L'histoire des harkis, c'est l'histoire d'une loyauté française et d'une fidélité déçue. Cette histoire, nous la regardons en face, avec ses ombres et ses lumières, avec la vérité comme exigence et la clarté comme guide. est l'objet et le sens du discours du Président de la République prononcé le 20 septembre dernier. À cette occasion, le chef de l'État a prolongé le chemin de la reconnaissance ouvert par Jacques Chirac et suivi par tous ses successeurs depuis Il a renouvelé la reconnaissance des manquements de la France et a rappelé la singularité de cette tragédie française. Il a souhaité aller plus loin- plus loin dans la reconnaissance, plus loin dans la réparation, plus loin dans la transmission mémorielle -, en annonçant l'inscription dans le marbre de nos lois de la reconnaissance et de la réparation à l'égard des harkis.

pour les harkis et leurs enfants, pour toutes les générations d'hommes et de femmes ayant subi la guerre d'Algérie, pour la mémoire nationale. C'est peu dire que nos discussions de ce jour sont attendues par les harkis, leurs associations, leurs enfants et leurs ayants droit. Nous savons, nous entendons les espérances et la soif de reconnaissance. L'examen en commission l'a très justement rappelé ; à ce titre, je tiens à saluer le travail mené par Mme la rapporteure et les membres de la commission.

de mes déplacements et lors de chaque cérémonie. Ce projet de loi s'inscrit dans le temps du pardon, ouvert par le chef de l'État. Il est celui de la reconnaissance par la Nation d'une profonde déchirure et d'une tragédie française, d'une page sombre de notre histoire. La France a tourné le dos à des combattants valeureux, qui l'avaient loyalement servie de 1954 à 1962. En cela, notre pays n'a été fidèle ni à son histoire ni à ses valeurs. Par ce texte, la France leur renouvelle sa gratitude ; car l'histoire des harkis est avant tout une histoire de soldats, d'hommes et de femmes servant sous le drapeau français. L'histoire des harkis, c'est aussi celle d'une tragédie : celle de femmes, d'hommes et d'enfants abandonnés sur leur terre natale ; celle de femmes, d'hommes et d'enfants rapatriés en métropole, déracinés et, pour certains, relégués. Pour toutes et tous, le 19 mars 1962, les accords d'Évian et l'application du cessez-le-feu ont été un tournant. Nous le savons : la vérité est cruelle. La France a tergiversé pour ouvrir ses portes aux harkis et à leurs familles. Pour ceux qui parvinrent à atteindre les rives du sud de la France, ce fut le début du déchirement et d'un douloureux exil, d'un temps d'incompréhension et d'incertitude. Ils attendaient l'hospitalité et la fraternité : ils ont souvent trouvé l'hostilité, voire l'arbitraire. Pour beaucoup, l'arrivée sur le sol métropolitain marqua le début des meurtrissures et de la marginalisation.

Près de la moitié d'entre eux a été reléguée, parfois durant des années, dans des camps et des hameaux de forestage. Vous le savez : ils y ont vécu dans des conditions de vie indignes. C'était en France ; c'était hier. Dans ces lieux, les harkis et leurs familles ont connu l'arbitraire, les barbelés, l'enfermement, le froid, les carences alimentaires, la promiscuité et l'absence d'intimité. Ils ont subi les brimades, les humiliations, les abus et les détournements de prestations ; autant de maux, autant de traumatismes. Je le rappelle, plusieurs milliers d'enfants ont été déscolarisés, mal accueillis et mal instruits. La France n'a pas été au rendez-vous de la plus belle des promesses républicaines, celle de l'école et de l'instruction. Ces lieux de bannissement ont meurtri, traumatisé et, parfois, tué. Cette situation, qui a duré, a été à juste titre ressentie et vécue comme une trahison. Conscient de ces souffrances et de leurs conséquences, notre pays, depuis plusieurs décennies et sous plusieurs gouvernements, a été aux côtés des harkis sur la voie de la justice et de la réparation. À cette fin, l'État a mis en place des dispositifs spécifiques. Il continue à les actualiser et poursuit le travail de mémoire. Toutes ces actions de mémoire, toutes ces mesures de réparation, nous les avons intensifiées depuis 2017. Conformément aux conclusions du rapport Ceaux, nous avons créé un dispositif de soutien pour la deuxième génération, pour les enfants de harkis ayant vécu dans les camps et hameaux de forestage. Nous aidons un nombre sans cesse croissant d'enfants de harkis à faire face à des dépenses d'insertion, de santé ou de logement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, par ce projet de loi, la République renouvelle la reconnaissance de ses manquements et couronne l'édifice de réparation. L'article 1 réaffirme la gratitude de la Nation à l'égard de tous les combattants qui ont servi la France entre 1954 et 1962. De plus, pour la première fois, la nation française reconnaît sa responsabilité dans les conditions indignes, précaires et attentatoires aux libertés pour l'accueil sur notre territoire de certains harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives, accompagnés de leurs familles. Nous ancrons dans la loi la journée nationale du 25 septembre et nous l'enrichissons d'un hommage aux compatriotes, aux officiers, aux particuliers et aux maires qui ont accompagné des harkis dans leur nouvelle vie sur les plans moral et matériel, pour les accueillir et les aider à s'intégrer. Ces femmes et ces hommes ont fait honneur à la France. Je me réjouis que nous trouvions les moyens de leur témoigner l'estime et la reconnaissance de la Nation. Ensuite, ce projet de loi précise le périmètre de la réparation des préjudices subis.

La réparation prend la forme d'une indemnisation forfaitaire et individualisée selon la durée du séjour dans les structures concernées. Les mesures de réparation accordées bénéficieront de règles d'exonération fiscale. Le texte instaure une commission nationale de reconnaissance et de réparation. Cette instance sera chargée de statuer sur les demandes de réparation après instruction par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre Parce que le travail de mémoire est essentiel, la commission mènera également une mission mémorielle pour recueillir, conserver et transmettre la mémoire des harkis. Enfin, ce projet de loi actualise les dispositifs préexistants et les renforce pour davantage d'équité. Il rend plus favorable le régime d'allocations viagères en supprimant les forclusions. telle disposition permet de rouvrir l'octroi de cette allocation aux conjoints survivants qui n'avaient pas présenté de demande dans le délai légal. Parallèlement, l'accès à l'allocation viagère est étendu aux personnes dont les conjoints décédés ont fixé leur domicile dans un pays de l'Union européenne et par la loi aux veuves des personnes « assimilées » aux membres des formations supplétives. Mesdames, messieurs les sénateurs, il n'est pas de meilleure reconnaissance que la connaissance. La transmission est donc essentielle et même prioritaire. L'histoire des harkis est trop méconnue des Français. Nous devons la faire connaître et favoriser son enseignement ; nous devons renforcer le travail mémoriel. Le souvenir des harkis est désormais rappelé sur les sites où ils ont vécu. Nous avons oeuvré pour reconnaître les mémoires les plus douloureuses ; je pense particulièrement au travail accompli autour des cimetières. La maison d'histoire et de mémoire d'Ongles, seul lieu de mémoire uniquement dédié à l'histoire des harkis, est soutenue par le ministère des armées. De même, un important travail d'archives et de collecte des témoignages a été déployé. Les expositions réalisées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont à la disposition de tous. Elles sont au coeur des actions menées dans les établissements scolaires. Bien sûr, les recueils mémoriels de la commission seront déterminants pour amplifier la transmission. Je connais l'attachement de la Haute Assemblée au monde combattant et son intérêt fort pour les enjeux de transmission, de reconnaissance et de réparation. Ainsi, ce projet de loi vous offre toute latitude pour renouveler l'hommage aux harkis, acter la reconnaissance de l'accueil indigne, ouvrir un nouveau chemin de la réparation et déterminer les conditions y ouvrant droit.

C'est pour la France une question de dignité et de fidélité. La République ne laissera pas l'injure raviver les douleurs du passé. Elle ne laissera pas l'abandon s'ajouter au sacrifice. Elle ne laissera pas l'oubli recouvrir la mort et la souffrance. » Par ces mots prononcés le 25 septembre 2001, le Président Jacques Chirac reconnaissait la responsabilité de la Nation dans l'abandon des harkis et des autres supplétifs qui avaient fait le choix de la France, au péril de leur vie. l'engagement des harkis, leur abandon, les traumatismes et les difficultés qu'ils ont subis, j'en ai reçu le témoignage en entendant, pour l'examen de ce projet de loi, des harkis et des membres de leurs familles. Leur parole est poignante, bouleversante, et leur histoire est celle de la France. Aux côtés de l'armée, la France a pu compter sur l'engagement de milliers de supplétifs d'origine algérienne : harkis, moghaznis, auxiliaires de la gendarmerie, groupes d'autodéfense, groupes mobiles de police rurale. S'y ajoutent plusieurs catégories de personnes assimilées aux membres des formations supplétives, à l'instar des agents de renseignements, des gardes champêtres ou des auxiliaires médico-sociaux des armées. À la fin de la guerre, le plan général de rapatriement du Gouvernement ne permet de rapatrier qu'une partie des anciens supplétifs, accompagnés de leur famille, dont la sécurité était menacée en Algérie. Nombre de ceux qui sont restés en Algérie, abandonnés, livrés à leur sort, considérés comme des traîtres, sont alors victimes d'exactions indescriptibles et assassinés malgré les engagements du Front Sur les 82 000 rapatriés d'origine algérienne qui sont arrivés en France, 42 000 anciens supplétifs et membres de leurs familles ont été accueillis dans des camps de transit et de reclassement, ainsi que dans des hameaux de forestage, où ils ont été engagés sur des chantiers d'aménagement de zones forestières. ces structures administrées par l'État ont subi des conditions de vie indignes et précaires : promiscuité, difficultés d'accès à la nourriture, brimades, humiliations, privations, déscolarisation des enfants, restrictions de circulation. le quotidien des harkis et de leurs familles est fait de souffrances et de traumatismes durables. Sous la responsabilité de l'État, ces structures, auxquelles il est difficile d'accoler le mot d'accueil, imposent des conditions de vie contraires aux lois et aux valeurs de la République. Après une révolte menée par les enfants de harkis, la fermeture administrative des derniers camps est décidée en conseil des ministres le 6 août 1975. Toutefois, nombre de familles de harkis y sont demeurées pendant plusieurs décennies, parfois jusqu'à aujourd'hui, notamment au camp de Bias. On ne peut le nier : depuis lors, de nombreuses mesures d'aide, de reconnaissance et d'indemnisation ont été déployées pour les anciens supplétifs et leurs ayants droit. Aides sociales à la réinstallation, indemnisation des biens perdus en Algérie, mesures de désendettement, aides au logement, possibilité de rachat de trimestres de retraite pour les enfants ayant séjourné dans les camps, emplois réservés dans l'administration : tous ces dispositifs ont bénéficié à des milliers d'anciens harkis et à leurs familles, en complément de l'aide sociale de droit commun. En parallèle, le devoir de reconnaissance et de mémoire envers les harkis s'est traduit depuis 2001 dans la parole présidentielle. Les Présidents Chirac, Sarkozy et Hollande ont successivement rendu hommage à l'engagement des harkis et reconnu que la République les avait abandonnés. Le 20 septembre dernier, le Président Macron a réaffirmé cette reconnaissance envers les harkis, en leur présentant, au nom de la Nation, une demande de pardon et en annonçant des mesures de reconnaissance et de réparation qui trouvent leur traduction dans le projet de loi que nous examinons aujourd'hui. La reconnaissance de la Nation, exprimée à l'article 1, recouvre deux aspects. D'une part, cet article réaffirme la reconnaissance de la Nation envers l'ensemble des supplétifs qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. Cette reconnaissance avait déjà été exprimée par la loi en 1994 et en 2005. Elle est complétée à l'article 1 par l'inscription dans la loi de la journée nationale d'hommage aux harkis, fixée au 25 septembre. D'autre part, l'article 1reconnaît la responsabilité de l'État du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire qui ont été réservées aux anciens supplétifs et à leurs familles hébergés dans des structures fermées où ils ont subi des conditions de vie précaires et des atteintes aux libertés individuelles, à savoir les camps de transit et les hameaux de forestage. Tirant la conséquence de cette responsabilité de l'État, l'État, l'article 2 institue un mécanisme de réparation financière en faveur des rapatriés ayant transité par un camp ou un hameau entre la publication des accords d'Évian, le 20 mars 1962, et la fin de l'année de la fermeture administrative des camps et des hameaux, le 31 décembre 1975. Pourront bénéficier de cette réparation les anciens supplétifs et les membres de leurs familles ayant séjourné dans l'une de ces structures entre 1962 et 1975. Seule la preuve du séjour sera à apporter par les demandeurs, le préjudice qu'ils ont subi dans ces structures étant présumé. Une somme forfaitaire, versée selon un barème fixé par décret, tiendra lieu de réparation. Le montant maximal devrait ainsi s'élever à 15 000 euros pour un séjour de 1962 à 1975, soit la somme au paiement de laquelle l'État a été condamné par le Conseil d'État en 2018 pour un séjour d'une durée comparable. La liste des structures concernées, fixée par décret, devrait être identique à celle des camps et hameaux retenus dans le cadre du fonds de solidarité envers les enfants de harkis créé à la La commission a précisé à l'article 1 qu'étaient concernées des structures de toute nature, afin que certaines prisons reconverties en lieux d'accueil pour rapatriés puissent également être comprises dans la liste des structures retenues. Le champ de la réparation prévue par le texte n'inclut pas les 40 000 rapatriés d'origine algérienne n'ayant pas séjourné dans ces structures, mais dans des cités urbaines, où les conditions de vie étaient également précaires, mais moins attentatoires aux libertés et droits fondamentaux. En effet, ces cités n'étaient pas soumises à un régime administratif dérogatoire du droit commun, contrairement aux structures fermées. On ne peut donc pas imputer à l'État la même responsabilité que celle qui est reconnue pour son administration des camps. Une telle extension créerait en outre une rupture d'égalité envers les autres personnes ayant séjourné dans ces cités au cours de la même période. Pour autant, une part importante des rapatriés ayant séjourné dans ces cités y ont été orientés après un passage en camp et pourront, à ce titre, bénéficier du droit à réparation. Les demandes de réparation seront soumises à une commission de reconnaissance et de réparation, créée par l'article 3, qui aura également la charge de recueillir et de transmettre la mémoire des harkis. L'histoire de ces citoyens français, la tragédie qu'ils ont vécue, la souffrance de leurs enfants et la douleur de leurs petits-enfants doivent être connues de tous. S'appuyant sur les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour l'instruction des dossiers, cette commission aura un rôle majeur, ce qui explique aussi la méfiance, voire les suspicions, qu'elle suscite. Sa création montre également que rien n'est figé. C'est la raison pour laquelle la commission des affaires sociales a souhaité renforcer les garanties de son indépendance. l'article 7, très attendu par la population harkie, lève plusieurs délais de forclusion applicables à l'allocation viagère, servie depuis 2016 aux conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens supplétifs ayant fixé leur domicile en France. La commission vous proposera, en accord avec le Gouvernement, d'étendre de quatre ans la période au titre de laquelle les veuves des anciens harkis pourront solliciter le bénéfice des arrérages de l'allocation viagère. Je remercie Mme la ministre d'avoir accepté notre demande, qui permettra la récupération des montants de l'allocation depuis sa date de création. Au total, si le texte qui nous est soumis comporte des avancées importantes pour améliorer la reconnaissance et la réparation envers les anciens supplétifs et les membres de leurs familles, ce projet de loi garde un goût d'inachevé. D'une part, je comprends parfaitement ceux qui considèrent qu'une somme de 15 000 euros n'est pas à la hauteur des souffrances endurées. Aucun montant ne permettrait de réparer intégralement un tel préjudice. D'autre part, le texte porte à titre principal sur un préjudice bien spécifique, subi par une partie des harkis et de leurs familles. reconnaissance ainsi proclamée n'est pas la reconnaissance due à l'ensemble des harkis. Le texte ne parvient donc pas pleinement à apaiser et à réunir la communauté harkie. « La douleur est énorme et si irrépressible qu'il est impossible de la combler » : tels sont les mots de l'historien Gilles Manceron, que j'ai auditionné ; je souscris pleinement à ces propos. C'est la raison pour laquelle la commission a considéré que, s'il contenait des avancées, ce projet de loi ne pouvait en aucun cas constituer un « solde de tout compte Notre discussion permettra- je le crois -de préciser que la réflexion doit se poursuivre sur l'opportunité d'instaurer de nouvelles mesures de reconnaissance et de réparation envers les harkis. La commission estime donc qu'adopter ce projet de loi permet de réaffirmer la reconnaissance de la Nation envers les harkis et de prévoir la réparation du préjudice subi par bon nombre d'entre eux.

Ce conflit terrible a fait des centaines de milliers de morts, dont 25 000 soldats français. La présence française en Algérie remontait à plus d'un siècle et les destins de nos populations s'étaient mêlés. La lutte qui a conduit à l'indépendance de notre ancienne colonie a revêtu une dimension de guerre civile, charriant les atrocités inhérentes à ces conflits particulièrement cruels. Des Algériens avaient pris fait et cause pour la France : les harkis, les moghaznis autres supplétifs. Au péril de leur vie, tout comme les soldats de métropole, mais sans bénéficier du même statut que ces forces régulières, ils ont servi notre pays.

hommage à la mémoire de ceux qui ont servi la France et qui ont payé cet engagement de leur vie et de celles des membres de leur famille. Nous ne devons pas les oublier. Parmi les 82 000

ceux qui se sont battus pour elle comme ses enfants. Ainsi a-t-elle manqué à son devoir. Le Gouvernement soumet aujourd'hui à notre examen un projet de loi dont l'objet est double. d'abord d'inscrire dans la loi la reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont servi la France et d'admettre que les personnes accueillies dans des conditions indignes ont subi un préjudice. Cette reconnaissance s'inscrit dans la lignée des déclarations que les Présidents de la République successifs ont pu faire. Elle n'en est pas moins importante, qu'il s'agisse des personnes concernées ou de notre travail de mémoire. ensuite, d'entreprendre la réparation du préjudice subi par ces populations, tâche délicate s'il en est, car la douleur et le temps perdu se convertissent mal en sommes d'argent.

d'impôts et de contributions sociales. Le dispositif prévu par le Gouvernement présente en outre l'avantage de la simplicité. L'indemnisation sera fonction du temps passé dans l'une des structures indignes qui furent destinées à les accueillir, et le préjudice sera présumé. dispensera les quelque 50 000 bénéficiaires potentiels de démontrer la réalité et l'étendue d'un dommage subi voilà maintenant un demi-siècle.

Par ailleurs, nous nous félicitons qu'une commission nationale indépendante soit constituée au sein de l'Office national des anciens combattants Elle aura pour mission spécifique de s'assurer que les démarches engagées sur le fondement de ce texte aboutissent. Elle aura aussi pour mission de contribuer à faire évoluer, le cas échéant, la liste des structures d'accueil au sein desquelles

de reconnaître les erreurs qu'elle a pu commettre et de tenter de les réparer. Tous les États ne font pas preuve de la même hauteur de vue. Nous tenons à saluer notre rapporteure, Marie-Pierre Richer, qui a accompli un excellent travail.

je tiens tout d'abord à remercier notre collègue Marie-Pierre Richer, rapporteure de ce texte, pour le travail appliqué et consciencieux qu'elle a mené. Comment ne pas penser, en cet instant, à ces hommes et à ces femmes qui, nous écoutant, attendent et espèrent ? Ils n'ont rien oublié de ces heures où l'indépendance de l'Algérie a soudain fait basculer plus d'un siècle d'histoire.

Ne rien oublier, c'est se souvenir que les harkis ont toujours cru en la France, s'acquittant de leur devoir envers elle dans les crises et les guerres. Des bords de la Marne au Mont-Cassin, le sang versé par les Algériens a souvent contribué à la destinée de notre pays. Ne rien oublier, c'est rappeler le courage qu'il fallut aux harkis pour faire ce choix au moment de l'indépendance de l'Algérie : le choix de la France. Ne rien oublier, enfin et surtout, c'est prendre conscience des conditions difficiles et même dramatiques dans lesquelles arrivèrent un million de femmes, d'enfants et d'hommes, contraints à un exil forcé, douloureux et sans retour.

je peux aisément vous dire combien ces lieux d'infortune furent précaires, honteux et misérables. Quel contraste terrible entre ce confinement au long cours et le prétendu confort moderne

métropolitaine. Certes, la France a mis en place des régimes d'indemnisation ; elle a aidé les veuves des anciens combattants et contribué à l'essor professionnel des enfants de harkis.

Au fond, mes chers collègues, donner plus à ceux qui ont moins pour compenser le déterminisme social et économique, n'est-ce pas, précisément, être fidèle à l'idéal républicain ?

toutes les victimes- je pense à celles qui arrivèrent ici, sur le sol métropolitain, par leurs propres moyens. Tel est d'ailleurs le sens d'un des amendements que j'ai déposés : il ne faut pas créer une injustice pour en réparer une autre.

Le Président de la République a demandé pardon aux combattants abandonnés. Mais que signifie cette demande de pardon si l'on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de ce que nous impose la vérité ?

furent les mots du Président de la République en septembre dernier. En 2016, François Hollande avait engagé cette reconnaissance de la responsabilité de la France dans le sort réservé aux harkis ; et en 2018 le Conseil d'État avait reconnu la responsabilité de l'État, condamné à indemniser un fils de harki en réparation du préjudice subi par celui-ci.

Comment le Gouvernement justifie-t-il de ne pas étendre cette reconnaissance et cette réparation à l'ensemble des harkis, y compris à celles et à ceux qui sont parvenus en métropole par leurs propres moyens après 1975 ?

ces seules structures. Comme l'indique notre rapporteure, « le champ de la reconnaissance n'inclut pas les 40 000 rapatriés d'origine algérienne n'ayant pas séjourné dans ces structures, mais dans des cités urbaines, où les conditions de vie ne se sont pas toujours avérées plus confortables, mais où ils n'étaient pas privés de la liberté de circulation

ont été jugés irrecevables pour raison financière. Nous demandons donc au Gouvernement d'assumer ses responsabilités en reprenant ces amendements à son compte. Puisqu'il le peut, il le doit ! Dans le même esprit, nous défendons la création d'une commission indépendante et diverse dans sa composition.

Oui, ce texte est incomplet et doit faire l'objet de modifications. Nous l'améliorerons donc ensemble ; je demande au Gouvernement de nous y aider. C'est notre travail d'oeuvrer en ce sens. Nous le devons bien aux harkis, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ainsi ce texte viendrait-il couronner une réflexion longue sur la place que notre pays n'a pas su leur octroyer. Mais il doit être bien plus que cela : il doit montrer notre volonté de nous confronter à notre histoire, si difficile soit-elle. En des temps où la réécriture du passé entache la démarche de vérité que nous nous devons à nous-mêmes, où les révisionnismes en tout genre tentent de gommer le travail de nos historiens, il m'apparaît judicieux de soutenir ce texte. Les harkis ont souffert des décisions de notre État. Leur abandon, péché originel, n'a pas été la dernière humiliation que la France leur a fait subir. Ils ont aussi été maltraités et oubliés, sans que tous ces préjudices soient reconnus

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 19 mars 1962 à midi, à midi, la guerre d'Algérie a pris fin avec l'entrée en vigueur des accords d'Évian. À la veille des célébrations du soixantième anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, le Président de la République a souhaité avancer vers la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la colonisation de l'Algérie de loi proclame la reconnaissance de la Nation envers les harkis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie. En prenant la décision d'abandonner à leur sort les harkis et leurs familles en Algérie, le gouvernement français de l'époque a trahi la parole donnée, condamnant ces femmes et ces hommes à des représailles sanglantes. Selon l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, 80 000 à 90 000 anciens supplétifs, épouses et enfants se sont réfugiés en France à compter du mois de mars 1962.

Aux privations de liberté et à la précarité des conditions de vie dans les camps et les hameaux de forestage se sont ajoutés les violences, les humiliations et le racisme. Ce projet de loi, qui prévoit d'accorder une réparation des préjudices subis au titre de l'indignité des conditions d'accueil sur le territoire français, constitue un progrès. Nous restons toutefois au milieu du gué en raison des critères d'indemnisation retenus. En effet, le processus de réparation se limite aux 42 000 harkis et membres de leurs familles qui sont passés par des structures comme les camps de transit et de reclassement.

ailleurs, en limitant la réparation aux harkis ayant vécu dans des structures d'accueil entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, le texte ne tient pas compte des familles qui y sont demeurées pendant de nombreuses années.

Enfin, le choix de verser une somme forfaitaire en fonction de la seule durée passée dans les camps pose question : il ne tient compte ni des circonstances ni des préjudices personnels endurés, parfois très lourds. Je pense notamment aux conjoints de personnes décédées, pour lesquelles la réparation devrait être plus importante, à rebours des critères envisagés dans l'étude d'impact. Au total, entre 40 000 et 50 000 harkis et membres de leurs familles sont exclus de toute réparation.

Néanmoins, en matière de mémoire, la reconnaissance ne saurait se réduire à la simple repentance et dépasse les dédommagements financiers ; elle exige de travailler sur les questions mémorielles dans un climat d'apaisement, de chaque côté, en Algérie comme en France. En effet, « si la mémoire divise, l'histoire peut rassembler », comme l'écrit l'historien Pierre Nora. Le rapport de Benjamin Stora préconise par exemple la constitution d'une commission « Mémoires et vérité chargée d'impulser des initiatives communes entre la France et l'Algérie. Pour ce faire, la France doit reconnaître sa responsabilité dans le massacre de Sétif, le 8 mai 1945,

La réconciliation de la France et de l'Algérie a été trop longtemps entravée par l'impossibilité de construire une mémoire commune entre nos deux pays. La France et les pays du Maghreb ont pourtant un rôle irremplaçable à jouer dans l'écriture de l'avenir du bassin méditerranéen.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens à saluer la qualité du travail de notre collègue rapporteure Marie-Pierre Richer sur un sujet certes passionnant, mais ô combien complexe. Le présent texte porte reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ayant transité par un camp ou un hameau de forestage entre 1962 et 1975. Cette page d'histoire est particulièrement tragique : plusieurs dizaines de milliers de harkis, considérés comme des traîtres, furent sauvagement assassinés sur le sol algérien. Militaires, civils, femmes, enfants ont été les victimes de ces terribles massacres. Parmi les 82 000 rapatriés d'origine algérienne ayant réussi à gagner la France, 42 000 personnes ont connu des conditions de vie indignes dans des camps de transit et des hameaux de forestage, où les anciens supplétifs étaient engagés pour travailler sur des chantiers d'aménagement de zones forestières. La souffrance, les atteintes aux libertés individuelles, la précarité, les humiliations, les privations et la déscolarisation des enfants ont marqué la vie de ces structures. Ce projet de loi s'inscrit donc dans une démarche de réparation des préjudices subis par ces personnes du fait de leurs conditions d'accueil sur le territoire français.

Il est essentiel de rendre hommage à l'engagement des harkis durant la guerre d'Algérie. Il est indispensable d'intensifier le soutien que la Nation leur apporte, ainsi qu'à leurs familles, afin d'améliorer leurs conditions de vie. Le principe d'une responsabilité de l'État envers les harkis a pris corps au fil des dernières décennies. Comme l'a rappelé notre collègue rapporteure, en complément de l'aide sociale de droit commun, des milliers d'anciens harkis et leurs familles ont pu bénéficier d'un grand nombre de mesures d'aide et de reconnaissance : aides sociales à la réinstallation, indemnisation des biens perdus en Algérie, mesures de désendettement, aides au logement, Par ailleurs, plusieurs mesures financières ont été prises depuis le 1 janvier 2017, par exemple la revalorisation de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère prévue en faveur des conjoints survivants de harkis. Ce texte instaure de nouvelles mesures de reconnaissance et de réparation. Il pose le principe de la responsabilité de la France dans l'indignité des conditions de vie qui ont été réservées à ces personnes sur son territoire. Le Gouvernement estime le nombre de bénéficiaires potentiels du dispositif à 50 000, pour un coût global de 302 millions d'euros. L'indemnité de réparation ne serait assujettie ni à l'impôt sur le revenu ni à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement. Les mesures d'aides sociales élargissent les conditions dans lesquelles peut être versée l'allocation viagère. Je salue la création d'une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et par les autres personnes rapatriées d'Algérie. Cette commission assurera la mission de recueil et de transmission de la mémoire ; elle aura un rôle décisionnel et de pilotage dans la procédure de demande de réparation. Aucun mot ne peut décrire le comportement de l'État à l'égard des harkis au lendemain de la guerre d'Algérie. Un sentiment d'abandon pèse toujours sur le coeur des survivants et sur celui de leurs descendants. Nous considérons que ces mesures ne peuvent en aucun cas constituer un « solde de tout compte » dans la reconnaissance due par la Nation aux harkis, qui ont participé au conflit au service de la France. Nous reconnaissons leurs souffrances et leurs sacrifices et tenons à rendre hommage à leurs familles.

Évidemment, la réalité est loin d'être satisfaisante. Évidemment, aucune mesure ne suffira jamais pour réparer toutes les violences, la souffrance, les atrocités subies par les harkis et par leurs familles. Évidemment, aucune indemnité financière ne peut aider à refermer les plaies. Certaines erreurs n'auraient tout simplement pas dû être commises par la France. Après plus de soixante ans, est-il encore possible de réparer l'irréparable ? Malgré le retard accumulé, ce texte représente une avancée et s'inscrit dans une trajectoire de réparation des blessures d'un passé toujours proche et vivant.

Parce qu'ils avaient servi la France, ils eurent le choix entre la mort et l'exil. Dans ces conditions, les harkis n'ont pas hésité à passer, quand ils l'ont pu, de l'autre côté de la Méditerranée, où l'horizon leur paraissait plus clair. Quelle déception ! La terre promise ne s'est pas révélée aussi accueillante qu'elle aurait dû l'être. Pour une partie d'entre eux, près de 42 000, le passage ou l'installation dans des camps de transit et de reclassement ou des hameaux de forestage a constitué une véritable relégation faite de souffrances et de légitime amertume. Dans ces camps qui, rappelons-le, étaient fermés, précarité, privations, déscolarisation et brimades étaient le lot quotidien des harkis- notre collègue rapporteure l'a très bien souligné. Il faut le dire : c'est l'indignité légalisée qui figurait au fronton obscur de ces structures, en lieu et place de la fraternité qui aurait dû y être prodiguée. Notre pays- patrie des droits de l'homme, dit-on souvent -a clairement raté, à cette époque, le rendez-vous de la compassion à l'égard de ceux qui croyaient en elle et qu'elle aurait dû accueillir avec plus de générosité. À Bias, en Lot-et-Garonne, à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, ou au Larzac, dans l'Aveyron, est-il compréhensible que de jeunes enfants aient longtemps vu la France des barbelés avant de connaître celle des libertés

loi, lequel institue un mécanisme de réparation financière en faveur des rapatriés ayant transité par un camp ou par un hameau de forestage entre 1962 et 1975. Nous approuvons également les articles renouvelant ou approfondissant la reconnaissance de la Nation à l'égard des harkis. la mesure relative à l'allocation viagère : la suppression de la forclusion permettra à des familles qui ignoraient leurs droits de les exercer. Toutefois, comme le souligne la commission, ce texte ne saurait constituer le solde de tout compte ». Une majorité des sénateurs de mon groupe aurait d'ailleurs souhaité étendre le bénéfice du dispositif de réparation à tous les harkis,

pour régler la situation des quelque vingt-cinq supplétifs de statut civil de droit commun dont le sort est régulièrement discuté au titre des projets de loi de finances. En attendant ces améliorations, le RDSE approuvera le projet de loi qui concrétise la demande de pardon formulée par le Président de la République.

et acceptant de l'être, résigné à ma singularité et à mes infirmités. Et je dois reconstruire une vérité, après avoir vécu toute ma vie dans une sorte de mensonge. C'est précisément ce que ressentent les harkis et leurs descendants, témoins et victimes d'une histoire coloniale douloureuse. Après l'enfer de la guerre d'Algérie, ceux qui ont combattu pour la France ont été abandonnés par elle. Ils ont été livrés à leur sort sur le sol algérien

sont glaçants. De telles conditions de vie ont emporté de graves conséquences sur l'état physique, psychique et psychologique de ces personnes. Les dommages matériels et moraux sont nombreux et irréversibles. Le temps du silence

En dehors d'une réparation pécuniaire, la reconnaissance solennelle des préjudices subis par les harkis et par leurs descendants est un tournant mémoriel dans l'histoire postcoloniale française. L'État ne peut se contenter de demi-mesures ou d'une loi incomplète. Il ne suffit plus de reconnaître ses torts ou de demander pardon, il est temps d'assumer pleinement ses actes. Pour ceux qui ont connu le pire de notre administration, pour ceux qui ont été privés de libertés fondamentales, pour ceux qui ont tout perdu pour la France, arrive enfin le temps de la vérité et de la cicatrisation. Ce texte est un premier pas : nous attendons la suite. À ce titre, je regrette que certains de nos amendements n'aient pas été jugés recevables. à vous remercier

Nous examinons un projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers l'ensemble des supplétifs qui ont servi la France en Algérie et que celle-ci a abandonnés. Ce texte reconnaît également- il faut nous en féliciter ! -la responsabilité de l'État français dans l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire réservées aux anciens supplétifs et à leurs familles, hébergées dans des structures fermées. Ce projet de loi s'inscrit dans la continuité des discours présidentiels, notamment celui de François Hollande, qui, pour la première fois en 2016, a reconnu explicitement la responsabilité des gouvernements français dans l'abandon des harkis, les massacres de ceux restés en Algérie et les conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France.

L'histoire des harkis, c'est l'histoire de la France, de notre Nation, qu'il nous faut regarder avec lucidité. C'est l'histoire de ces Français, nés en Algérie, qui ont été recrutés pour appuyer l'armée française durant la guerre d'Algérie.

L'histoire des harkis est aussi celle d'un abandon. À la fin de la guerre, le gouvernement français ordonne à l'armée de désarmer les harkis et de limiter strictement leur rapatriement : il a, de fait, laissé sur place Seuls sont rapatriés les Français d'origine européenne et une partie des anciens supplétifs, dont la sécurité est menacée en Algérie. Les anciens harkis, considérés comme des traîtres en Algérie, sont victimes d'exactions et de massacres sur le sol algérien. abandon se poursuit sur le sol français : sont frappés ceux qui ont réussi à être rapatriés, souvent grâce à la désobéissance de certains officiers français, hommes d'honneur qui, faisant fi des ordres donnés, ont organisé eux-mêmes le rapatriement de leur harka.

soumis à un régime dérogatoire du droit commun, isolés à plusieurs kilomètres des villages, devant subir un couvre-feu et le contrôle de leurs déplacements. Ils connurent des conditions d'hygiène déplorables et subirent le manque de scolarisation de leurs enfants.

En effet, le champ de la reconnaissance n'inclut pas les 40 000 personnes n'ayant pas séjourné dans ces structures, alors que leurs conditions de vie ne se sont pas toujours révélées plus dignes. De plus, au-delà des sommes allouées, le système de forfait n'est pas à la hauteur des préjudices dont furent victimes les harkis et leurs familles. Il n'est en aucun cas une reconnaissance par la Nation des violences vécues. Un tel forfait, c'est l'acceptation d'un préjudice sans la reconnaissance de la culpabilité. Tous les anciens harkis et leurs familles méritent que leur histoire et leurs souffrances soient entendues et bénéficient d'une réparation individuelle, fondée sur ce que chacun d'entre eux a réellement subi.

qui participe de notre richesse, celle de la réconciliation nationale et du vivre ensemble. Ce texte constitue une avancée, mais il ne saurait être un solde de

soit délaissés sur leur terre natale, en proie aux exactions et aux massacres, soit rapatriés en métropole, coupés de leurs racines et relégués dans des cités urbaines, des camps ou des hameaux de forestage. Dans ces camps et ces hameaux de forestage, où certains ont passé des années, ces personnes ont connu l'abandon, l'enfermement et la survie dans des conditions particulièrement précaires et indignes. Leur vie était dominée par le rationnement, la faim, le froid, la promiscuité, la maladie, l'exclusion, les privations privations de libertés, l'arbitraire et le racisme, au mépris des valeurs qui fondent notre République, au mépris du droit et de toute justice. Ces souffrances se sont transformées en traumatismes durables, que nous savons difficiles à apaiser complètement, soixante ans plus tard. C'est pourquoi, le 20 septembre 2021, le Président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole pour demander pardon au nom de la France. Pour réparer cette faute de l'État que fut l'indignité de ces conditions d'accueil et de séjour sur le territoire national, dans ces camps et hameaux de forestage, il a reconnu la nécessité d'inscrire dans le marbre de la loi la responsabilité de l'État d'indemniser et de rendre justice.

: il acte la création d'un mécanisme de réparation des préjudices subis par ces personnes, leurs conjoints et leurs enfants dans les structures visées.

La commission nationale de reconnaissance et de réparation, créée par l'article 3, sera au coeur de ce dispositif. Elle a gagné à l'Assemblée nationale la faculté « de proposer des évolutions de la liste des lieux » dans lesquels il est nécessaire d'avoir séjourné pour bénéficier du mécanisme de réparation. Cette lui confère les moyens d'être une entité active capable de détecter les angles morts et de faire évoluer le mécanisme de réparation. Sa mission mémorielle est tout aussi déterminante : en recueillant de nouveaux témoignages, elle sera en mesure d'aider à transmettre aux jeunes générations la mémoire la plus précise possible, pour que rien ne soit oublié. Enfin, c'est un véritable soulagement que l'article 7 vienne supprimer les irritants relatifs à l'allocation viagère, qui empêchaient injustement plusieurs veuves d'y accéder. Félicitations, madame la rapporteure ! Notre groupe tient à vous remercier de votre travail minutieux et des précisions essentielles que vous avez apportées à ce texte en commission. Je pense notamment à votre amendement tendant à préciser que la responsabilité de l'État concernera des structures « de toute nature » ayant fait subir à leurs résidents des conditions indignes et attentatoires à leurs libertés, ce qui ouvre la voie à l'inclusion de certaines prisons reconverties en lieux d'accueil pour les harkis, pour l'heure encore mal identifiées.

désormais sans ambages -, à la demande de la commission, l'ONACVG sollicite systématiquement de tout service de l'État, collectivité publique ou organisme gestionnaire de prestations sociales la communication de tout renseignement utile à l'exercice de ses missions.

Le premier tend à préciser les conditions de désignation des membres qui siégeront au sein de la commission en confiant cette prérogative au Premier ministre, sur proposition des autorités compétentes. Notre préoccupation,

Parce que ces hommes courageux avaient servi sous le drapeau français, ils furent, avec leurs familles, victimes de représailles après le cessez-le-feu, car privés de la protection de la France. Pour survivre et ne pas subir le sort de près de 100 000 de leurs compatriotes, massacrés par l'organisation terroriste du FLN, ils furent condamnés à un exil précipité. Bravo ! Oui, en Algérie, la France a abandonné une partie de ses propres soldats.

Je veux simplement croire que le Président Macron se repent- oui, se repent ! -des propos ignobles qu'il a tenus en 2017 à Alger, en qualifiant la présence française en Algérie de crime contre l'humanité.

Certains ont voulu croire en la parole du chef de l'État. Leur espoir était immense, pour qu'enfin soit reconnue l'indignité de leurs conditions d'accueils. Malheureusement, cet espoir est déçu. n'a jamais dit que près de la moitié des harkis seraient exclus de la réparation. Leur seul tort est de ne pas avoir vécu entourés de barbelés. En hiérarchisant la souffrance, vous bafouez leur honneur et leur loyauté ; en les condamnant à leur sort, vous créez une défiance qu'il vous faudra

lorsque est portée à l'égard d'un harki une injure ou une diffamation ; rien de l'abrogation de la journée du 19 mars, date funeste qui, par l'ampleur des massacres commis, n'a pas empêché le sang de couler, bien au contraire. Les harkis ont eu le

ans après les faits, des extrémistes se détournent de notre pays selon une logique victimaire anti-France, comment ne pas ériger en héros et en exemples ces musulmans qui ont combattu pour la France ?

Les harkis ont montré la voie dans cet inconnu permanent de l'avenir qui, un jour, devient histoire. J'en appelle à votre sens du devoir pour que les harkis, qui ne demandent pas la charité, ne subissent pas une énième trahison, eux qui avaient choisi de se ranger du côté de la France. Tout doit commencer par la vérité tout doit finir par la justice.

Mes premiers mots iront aux harkis, à leurs familles, aux blessés, aux âmes écorchées, aux morts. Je tiens à rendre hommage eux, où qu'ils aient vécu, avant ou après 1975. Les auditions du Sénat et de l'Assemblée nationale ont fait ressurgir en moi, fille de pieds-noirs, nombre de souvenirs, de témoignages, d'histoires et de visages. Ils m'ont laissée muette face à la douleur vécue, face à la blessure de l'histoire, face à la vérité criante qui domine chacun de ces témoignages : le cessez-le-feu n'en était pas un ; la guerre a continué ; les accords de paix cachaient une paix bâclée. bâclée. Au sommet de l'État français régnait la peur- peur laissée par le souvenir de la guerre d'Indochine, peur de s'enliser dans une guerre interminable. La peur a mené à la précipitation. Doublée d'un manque de considération, elle a rendu l'État, la France, lâche.

Les Présidents Hollande et Sarkozy ont eu des mots forts pour les harkis ; le Président Macron aussi. Ils savent que les harkis n'oublient pas et que jamais au grand jamais ils n'accepteront un énième abandon, une énième lâcheté. Les harkis honorent la Nation et le peuple français par leur courage, par leur patriotisme, par leur amour de la France. Ils donnent une chance à l'État de sortir d'un silence sournois, d'une pudeur qui entache l'esprit français. N'oublions pas qu'il s'agit d'une réparation par la France, pour la France, pour son unité. Voilà pourquoi l'injure faite aux harkis est une injure faite à la Nation. Déclassifions les archives, continuons les auditions : les préjudices ne sont pas encore tous établis. Madame la ministre, je forme le voeu que l'office national indépendant, création de ce gouvernement,

Aux associations de harkis, je veux dire que la loi peut paraître froide, mais qu'elle n'est jamais une fin en soi. N'ayez pas peur, car le chemin ne s'arrête pas là. Ce gouvernement instaure, le 25 septembre, la journée nationale d'hommage aux harkis. Chaque année, mesdames, messieurs les harkis, la République vous entendra. Chaque année, nous essaierons ensemble de faire un pas de plus vers l'apaisement. Comme l'indiquait ma collègue Jocelyne Guidez, les membres du groupe Union Centriste voteront en faveur de ce texte. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous réunit aujourd'hui se doit de répondre enfin aux aspirations de milliers de nos compatriotes : les harkis et leurs familles. Les harkis servaient dans les forces armées françaises. Ils étaient moghaznis, tirailleurs, spahis, membres des forces régulières, des groupes mobiles de sécurité, des groupes d'autodéfense et des sections administratives. Ils furent 200 000. Nous leur devons remerciements et reconnaissance. Ils ont risqué leur vie pour une patrie qui était et qui demeure la leur : la France. Pourtant, après la proclamation du cessez-le-feu

ne furent ni protégés ni rapatriés, mais abandonnés à leur triste sort. Alors, il fallut le courage et la parole de nombreux militaires français, au nom de la fraternité d'armes, pour assurer le rapatriement en France de près de 90 000 soldats harkis et de leurs familles.

Des enfants morts de faim et de froid, enterrés sans sépulture, d'autres déscolarisés, des femmes violentées et humiliées, parfois même violées, l'internement en cas de rébellion, l'insalubrité et la promiscuité au quotidien, la spoliation des maigres revenus par les chefs de camp : chacun peut imaginer les conséquences de telles épreuves

qu'ils furent rejetés de l'autre côté de la Méditerranée et mal acceptés ici même, dans leur pays, la France. Les harkis durent attendre douze années après la fin de la guerre d'Algérie pour obtenir le statut, pourtant légitime, d'anciens combattants.

n'est pas se repentir ; c'est admettre l'expression de la douleur vécue. Il nous faut être respectueux. Le respect est la marque à laquelle on reconnaît l'humanité et c'est toujours l'honneur d'un pays. Madame la ministre, les associations de harkis attendaient beaucoup de ce projet de loi, né de la volonté présidentielle, le 20 septembre dernier, à l'Élysée- j'y étais. Elles sont déçues et parfois même en colère. Il n'y a pas eu de concertation et ce texte présente

c'est avec beaucoup d'émotion et de gravité que nous abordons ce projet de loi et, avant tout, je tiens à remercier notre rapporteure, Marie-Pierre Richer, de son travail et de son sens de l'écoute. Cette reconnaissance de la Nation envers les harkis découle d'un long processus, engagé dès 2001 par le Président Jacques Chirac et qu'il convient de poursuivre.

À la fin de cette guerre, la France a rapatrié une partie des anciens supplétifs, accompagnés de leurs familles, dont la sécurité était désormais menacée sur la terre qui les avait vus naître. Sur ce même sol, plusieurs dizaines de milliers de harkis furent assassinés.

Parmi les harkis ayant pu être rapatriés, 82 000 étaient d'origine algérienne, dont 42 000 furent accueillis dans des conditions indignes se traduisant par des atteintes aux libertés individuelles, une forte précarité, des brimades ou encore la non-scolarisation des enfants.

Nous sommes nombreux, au sein de cet hémicycle, à déplorer le communautarisme. Oui, notre République, riche de sa diversité, nourrit l'ambition humaniste de ne faire qu'un

Nous saluons cette reconnaissance, très attendue par les anciens harkis. L'article reconnaît également la responsabilité de la Nation à l'égard de ces personnes pour l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans les camps et hameaux de forestage, entre 1962 et 1975.

Nous en sommes convaincus, un droit à réparation individuelle et une reconnaissance non discriminatoire seront sources d'apaisement.

et accueilli ces citoyens français, dont le seul tort aura été d'aimer la France, de la servir et de la défendre. Le patriotisme des harkis a été bien mal récompensé : la mère patrie pour laquelle ils se sont engagés au péril de leur vie les a abandonnés.

en lieu et place des armes qui leur servaient à défendre la France et qui leur ont été retirées, de sorte qu'ils ont été livrés aux représailles. J'ai écouté le silence assourdissant de ces hommes et de ces femmes qui, par pudeur ou par épuisement, ne pouvaient ou ne voulaient plus évoquer les exactions et les humiliations endurées.

les hameaux de forestage de mon département, à Saint-Pons-de-Thomières, à Lodève et à Avène, et les centres de transit de ma région, à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, à La Cavalerie en Aveyron et à Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard.

parole est à M. Olivier Paccaud, sur l'article. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il est dans l'histoire de France bien des heures glorieuses, mais il est aussi des pages plus sombres, enfouies sous un oubli gêné. C'est le cas de la guerre d'Algérie, dont notre mémoire collective a tant de mal à s'emparer. Les plaies ne sont pas cicatrisées, peut-être parce que ces « tristes événements », comme on les a longtemps faussement appelés, ne sont pas si lointains ; peut-être aussi parce que notre nation souffre de n'avoir pas su trouver une issue moins sanglante et cruelle à ce conflit. Certes, rien n'était simple. Entre l'attachement des pieds-noirs au sol d'Afrique, la détermination des indépendantistes algériens et l'impatience de la métropole à sortir de ce bourbier, où tant d'appelés laissèrent leur vie ou leur jeunesse, l'Algérie fut un récif tranchant sur lequel se brisèrent plusieurs gouvernements et même une République. À la fois guerre civile et guerre d'indépendance, la tragédie algérienne est une page de ce passé qui ne passe pas. S'il était difficile, voire impossible, de résister au vaste mouvement de décolonisation, et de l'Organisation armée secrète (OAS) ne cessait de fortifier ce nid de scorpions, le sort réservé aux harkis à la fin du conflit n'est à l'honneur ni de la France ni de l'Algérie. Ces citoyens français fidèles à la France furent, après les accords d'Évian, doublement persécutés. Abandonnés d'un côté, pourchassés de l'autre, ils périrent par milliers. Pour ceux qui eurent la chance de traverser la Méditerranée et de rallier la France, l'accueil, souvent dans des camps ou des structures de fortune, ne fut pas toujours chaleureux. Injustement oubliés et négligés, nos amis harkis méritent l'hommage de la nation française tout entière, car c'est leur nation. Leur sacrifice et leur amour de la France ont longtemps été ignorés. Il est temps de le reconnaître. Il est temps de rendre aux harkis, à ces braves et à leurs descendants, ce que la France leur doit. Ce texte constitue une avancée réelle, mais perfectible. À nous de l'améliorer pour que la France puisse enfin regarder ses fils harkis droit dans les yeux.

on ne nous prend pas en considération, nous ne sommes sur aucune liste. » Conjointement avec le maire de la commune, M. Laurent Baude, avec les harkis du Loiret et leurs représentants, je vous le demande

Dans leur immense majorité, ces anciens supplétifs réfugiés en France métropolitaine sont juridiquement redevenus français par la procédure de déclaration recognitive qui leur a été ouverte jusqu'en 1967 par l'ordonnance du 21 juillet 1962. L'ambition de ce projet de loi étant de « reconnaître la responsabilité de la France du fait des conditions indignes de l'accueil des personnes anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles, rapatriées d'Algérie, sur son territoire après les accords d'Évian et de réparer les préjudices subis par ces personnes résultant de leurs conditions de vie, particulièrement précaires, dans les structures de transit et d'hébergement où ils ont été cantonnés », il convient de nommer justement les événements et les personnes impliquées. Je rappelle que les Je rappelle que les harkis étaient des militaires français et qu'ils ont versé leur sang lors de plusieurs conflits, en France métropolitaine ou ailleurs.

Ils ont perdu la nationalité française lors de la conclusion des accords d'Évian, mais l'ont recouvrée progressivement grâce à l'ordonnance du 21 juillet 1962. Cet épisode fâcheux a été vécu par les intéressés comme une marque d'indignité infligée par la mère patrie. Plus récemment, certains d'entre eux me disaient qu'ils l'avaient ressenti comme une déchéance de nationalité, comme une infamie de plus. Il convient de proclamer dans la loi, une bonne fois pour toutes, que les harkis ont été

Cet amendement vise à entériner la qualité de Français des harkis qui ont combattu en Algérie. Comme l'ont dit les orateurs précédents, les harkis se sont battus pour la France et ils étaient bel et bien français avant de perdre cette nationalité

du 19 mars 1962 comme « la fin des combats, le soulagement pour beaucoup, l'angoisse pour tant d'autres, le début du calvaire pour les harkis, la cruauté des représailles, l'exil ou la mort ». En somme, les harkis ont eu le choix entre la valise et le cercueil. Si la France ne saurait reconnaître la responsabilité de massacres qu'elle n'a pas commis,

aux autres citoyens et enfants de la République. Élargir la reconnaissance de la faute de la France à l'endroit de la deuxième génération, passée par les camps, hameaux de forestage et foyers, particulièrement quand l'État a failli à son devoir de scolarisation des enfants, constituerait une avancée sans précédent, que le Président de la République a d'ailleurs appelée de ses voeux dans son discours du 20 Ensuite, il s'agit de recueillir les témoignages et de réparer [les préjudices] pour la deuxième génération qui a eu à vivre les camps, qui a eu à vivre les hameaux de forestage ou les foyers dans des conditions de vie indignes et l'absence d'accès à l'école pour les enfants. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence les paroles prononcées par le Président de la République et ce texte de loi. Il s'agit également de reconnaître que ceux qui ont été relégués dans les structures d'hébergement ou de transit ont subi divers préjudices, allant de la privation de liberté à la spoliation. L'amendement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

fidèles à l'histoire des harkis. Ces derniers ont été abandonnés, désarmés par la France, laissés à leur triste sort face aux actes barbares du FLN. Tel est donc l'objet de cet amendement : reconnaître la responsabilité de la France, non seulement dans les conditions d'accueil des harkis, mais également dans leur abandon.

Cet amendement vise à éviter toute discrimination envers la communauté harkie, induite par une distinction fondée, dans la rédaction actuelle de l'article 1, sur les conditions d'accueil et d'hébergement sur le territoire français. français. Si ce projet de loi cible assez bien la reconnaissance des préjudices subis lors de l'accueil des harkis en métropole, il est dommageable de distinguer les structures ouvertes et fermées.

créée pour la circonstance à l'article 3, pourra instruire les demandes de reconnaissance et de réparation grâce à une enveloppe financière dédiée, annuelle et normée. Elle devra examiner toutes les formes de logement ayant abouti à une relégation.

Tous les supplétifs de l'armée française n'ont pas eu le choix entre partir en France ou rester en Algérie. Certains d'entre eux ont réussi à gagner l'Hexagone plusieurs années après le cessez-le-feu à leur arrivée, qu'ont-ils trouvé ? Rejet, misère et humiliation ! Il ne faut en aucun cas les exclure du texte et les priver de leur droit à la réparation. Cet amendement vise à réécrire le deuxième alinéa l'article 1

voire parfois dans l'hostilité. Ils ont de fait subi un préjudice. Circonscrire ce projet de loi à l'espace déterminé des structures de toute nature exclura, en violation du principe constitutionnel d'égalité des citoyens, des harkis qui ne sont pas passés par ces structures, mais qui seraient pourtant éligibles à une reconnaissance du préjudice subi du fait de leur statut.

Sur ce sujet, je serai clair : il s'agit de réparer d'abord pour la première génération et de pouvoir revaloriser les allocations pour les anciens combattants et leurs veuves, c'est un devoir. » Il poursuivait Ensuite, il s'agit de recueillir les témoignages et de réparer [les préjudices] pour la deuxième génération qui a eu à vivre les camps, qui a eu à vivre les hameaux de forestage ou les foyers dans des conditions de vie indignes et l'absence d'accès à l'école pour les enfants.

Cet amendement vise donc à ce que les traumatismes et les préjudices subis par les enfants accueillis dans ces conditions indignes soient reconnus et inscrits dans la loi. En résumé, les discours, c'est bien ;

Il prévoit ensuite de reconnaître la responsabilité de la Nation du fait de l'indignité des conditions d'accueil subies par certains harkis et leurs familles hébergés dans des structures telles que des camps et des hameaux de forestage- nous l'avons tous évoqué lors de la Rappelons que la reconnaissance de la Nation envers les harkis est déjà exprimée dans deux lois toujours en vigueur : celle du 11 juin 1994 et celle du 23 février 2005. Je regrouperai les amendements par thème, plusieurs d'entre eux ayant des objets analogues.

tous les supplétifs n'étaient pas français : certains Marocains et Tunisiens résidant en Algérie ont servi dans les harkas. Concernant les autres supplétifs, je tiens à être parfaitement claire : nul ne remet en cause leur qualité de citoyen français, qui a motivé leur engagement au service de la France. Je précise qu'aux termes de l'ordonnance du 21 juillet 1962, les supplétifs de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1 janvier 1963, sauf si, établis en France, ils ont souscrit avant le 22 mars 1967 une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Il ne me semble pas nécessaire d'inscrire cette précision dans la loi.

Si je souscris pleinement à l'intention des auteurs, je souligne que le gouvernement de l'époque n'a pas donné l'ordre de ne pas rapatrier les supplétifs, mais de limiter les arrivées au strict cadre du plan général de rapatriement. Rappelons également que le FLN s'était engagé à assurer leur sécurité après les accords d'Évian.

Les amendements n 4 rectifié et 44 tendent à mentionner la perte de chance subie par les harkis et leurs enfants. Ces amendements sont satisfaits, car le présent texte reconnaît déjà l'indignité des conditions d'accueil

La perte de chance subie par les enfants de harkis est prise en compte à la fois par ce texte et par les dispositifs d'aide existants, qui, je le rappelle, s'ajoutent à l'aide sociale

Les amendements n 43 et 33 rectifié tendent à adjoindre aux anciens supplétifs rapatriés d'Algérie ceux qui sont arrivés en France par leurs propres moyens. Or le terme « rapatriés » inclut tous les anciens supplétifs ayant servi en Algérie et s'étant installés en France, quel qu'ait été leur moyen de gagner le territoire national. Ainsi, toutes ces personnes et les membres de leur famille seront éligibles au droit à réparation, à la seule condition d'avoir séjourné dans un camp ou dans un hameau de forestage- c'est là le

Les amendements n 41, 42 et 15 rectifié visent, sous des rédactions différentes, à étendre le champ de la responsabilité de l'État à l'ensemble des harkis et de leurs familles en supprimant le critère de séjour dans des camps ou hameaux ou en élargissant ce critère à des structures « fermées ou ouvertes ». Je comprends parfaitement l'intention de leurs auteurs : il est certain que les harkis et leurs familles ont connu des conditions de vie précaires, qu'ils aient été ou non hébergés dans des camps. pourquoi l'alinéa 1 reconnaît leur engagement et leur abandon. En revanche, l'alinéa 2 cible une responsabilité de l'État pour un préjudice particulier, né des conditions d'accueil indignes et privatives de liberté subies dans les camps et hameaux, alors que ces structures étaient sous la responsabilité de l'État. Il y a là une faute imputable à l'État, que l'on ne peut pas étendre aux conditions de vie hors de ces camps. Voilà pourquoi le droit à réparation, prévu à l'article 2, ne pourrait par exemple pas être étendu à l'accueil dans des cités urbaines, lesquelles n'étaient pas soumises à un régime administratif dérogatoire du droit commun, contrairement aux structures fermées.

les graves atteintes aux droits et libertés subies par les harkis dans ces structures ainsi que la précarité de leurs conditions de vie. Nul ne peut en douter. Toutefois, le présent texte indique déjà que les conditions d'accueil étaient indignes, qu'elles ont été marquées par une précarité par des privations et atteintes aux libertés individuelles et aux droits fondamentaux. Ces termes me semblent suffisamment précis pour englober la diversité des conditions de vie subies dans ces structures- les camps, les hameaux ou les prisons reconverties.

En mai 1962, trois instructions de Pierre Messmer, ministre des armées, Louis Joxe, ministre des affaires algériennes, et Roger Frey, ministre de l'intérieur, ont rappelé l'interdiction des rapatriements hors de ce plan ; et, en septembre 1962, Georges Pompidou a décidé de l'accueil des harkis.

que nous voulons réparer avec ce projet de loi, comme s'y est engagé le Président de la République dans son discours du 20 septembre 2021.

Un oubli volontaire, conscient et assumé constituerait une insulte à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie à la France.

ils ont été loyaux envers la France : c'est pour cela qu'ils ont été stigmatisés, pourchassés et exterminés par les tueurs du FLN. Au nom de la vérité, au nom de la fidélité des harkis à la France, exauçons la volonté des descendants de ces braves. Rendons-leur justice en leur reconnaissant pour toujours cette citoyenneté française

pour tous les représentants du monde combattant, toutes les associations patriotiques et de mémoire, tous les porte-drapeaux, pour qui nous avons aussi beaucoup de respect et de reconnaissance, ce terme

Le samedi 25 septembre 2021, les harkis ont été doublement honorés dans mon département de la Drôme, le matin par une cérémonie au carré militaire de Valence, l'après-midi lors de l'inauguration d'une plaque commémorative au hameau de forestage de Beaurières, commune voisine de la mienne.

à vous citer les mots de Rekia Danet, arrivée enfant à Beaurières, qui décrit ainsi son hébergement : « On est arrivés fin 1962 : c'était l'hiver ; nous étions logés dans des tentes meublées avec de gros poêles à bois, des lits en fer et des tables de l'armée. « Quelques jours plus tard, il s'est mis à neiger neige nous arrivait aux genoux et ce n'était pas évident, car il fallait prendre le chemin de l'école, distante de trois kilomètres. Ma petite soeur, en voyant la neige, a dit à ma mère que c'était comme du sable mais que c'était froid.

communes environnantes, la solidarité s'est exercée sous la houlette d'André Reynaud, maire du village, qui n'hésitait pas à faire le tour des maisons et des commerces pour que chacun aide à porter vêtements et nourriture. Je me félicite que, lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, l'article 1 ait étendu la journée nationale d'hommage aux harkis à toutes les personnes qui leur ont porté secours et assistance. Ces dernières font honneur à la République, là où malheureusement l'État a failli. À Beaurières, les enfants étaient scolarisés ensemble au sein de l'école de la République, dans deux classes supplémentaires créées grâce à l'installation de préfabriqués dans la cour. Élisabeth et Pascal Reynaud, les enfants du maire, nous rappellent régulièrement qu'ils étaient tous assis sur les mêmes bancs et qu'ils jouaient ensemble sans distinction.

Je souhaiterais que ce texte permette à la République française de reconnaître la barbarie et l'ampleur des massacres commis après le 19 mars, notamment ceux de la rue d'Isly ou ceux d'Oran, le 5 juillet, et de parler des disparus

Jean-Jacques Jordi a déclaré : « De 1957 jusqu'aux accords d'Évian, il y a eu à peu près 330 disparus civils. On pouvait s'attendre à ce qu'après les accords d'Évian ce chiffre baisse. entre les accords d'Évian et la date de l'indépendance, le 5 juillet 1962, c'est-à-dire en quelques semaines, il y en a eu plus de 600, donc deux fois plus en quatre mois qu'en six ans de guerre. Je tiens à vous parler d'un autre événement extrêmement important : la fusillade de la rue d'Isly, cette fusillade unilatérale qui a duré douze minutes. La France n'a pas respecté le cessez-le-feu : le bilan officiel fut de 49 morts et 200 blessés toutes les victimes furent des civils, on ne déplora pas un mort chez les militaires. Les civils n'ont pas pu enterrer leurs morts dignement ; les obsèques religieuses ont été interdites ; les corps furent convoyés directement au cimetière par camions militaires au jour et à l'heure choisis par les autorités.

Personne n'en disconvient, mais il est juste de rappeler que des familles de harkis ont été victimes de représailles, d'exécutions sommaires et de sévices. Ces personnes n'étaient pas engagées dans l'armée française

non seulement des sacrifices qu'ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France, mais également des sévices qu'ils ont subis pour cette même raison. Il s'agit là d'une proposition pertinente. Il est indéniable que des milliers d'anciens supplétifs ont subi des persécutions et des massacres en raison de leur soutien

Ce que la loi a fait, la loi peut le défaire- je dirais même, doit le défaire. Le 6 décembre 2012,

Pour qu'une commémoration soit commune, il faut que la date célébrée soit acceptée par tous. Or chacun sait qu'il n'en est rien, le 19 mars reste au coeur d'un débat douloureux. Jacques Chirac, qui avait été sous-lieutenant durant ce conflit, choisit avec discernement une autre date d'anniversaire, celle du 5 décembre. Puis, il y eut le 25 septembre, une date qui apaise. Même François Mitterrand estimait la date du 19 mars, car « il y aurait confusion dans la mémoire de notre peuple. Ce n'est pas l'acte diplomatique rendu à l'époque qui pourrait s'identifier à ce qui pourrait apparaître comme un grand moment de notre histoire, d'autant plus que la guerre a continué, que d'autres victimes ont été comptées

de la date du 19 mars, celle-ci marque l'entrée en vigueur de funestes accords d'Évian, qui n'ont jamais signifié la fin des combats et des exactions. Après cette date, de sinistre mémoire, des milliers de harkis et de pieds-noirs ont perdu la vie dans des assassinats et des massacres, comme ceux comme ceux de la rue d'Isly et du 5 juillet à Oran. Commémorer les accords d'Évian, c'est commémorer l'abandon et la douleur subie par ceux qui se battaient pour la France. Si la France souhaite honorer la mémoire des harkis, qui l'ont choisie

Le présent amendement vise donc à abroger la loi de M. Hollande du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir

surtout l'objet de ces amendements, niant la responsabilité de l'Organisation armée secrète (OAS) dans la tuerie de la rue d'Isly, qui est inacceptable. Les historiens ont reconnu la responsabilité des activistes d'extrême droite de l'OAS dans la fusillade du 26 mars 1962, ayant entraîné le décès

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera contre ces amendements identiques, dont les auteurs revisitent et réécrivent l'histoire de la guerre d'Algérie, au mépris des milliers de victimes qu'elle a suscitées.

au premier chef, comme tous les Français des trois départements d'Algérie, par ce qui s'est passé après le 19 mars. C'est la raison pour laquelle nous demandons depuis des années, avec un certain nombre de mes collègues, dont Philippe Tabarot, que cette date soit revue.